J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 21 voix pour, 3 voix contre et 7 bulletins blancs -à la nomination de M. Julien Boucher aux fonctions de directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ! Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires, présentée par Mme Marie-Pierre Monier et plusieurs de ses collègues et de la proposition de loi tendant à abroger la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée

dispositions étaient sans doute trop éloignées du coeur du texte initial : c'est en tout cas ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel, estimant que vingt-trois articles introduits en cours d'examen par les parlementaires n'avaient pas de lien, même indirect, avec le texte. Pour autant, nombre de ces nombre de ces dispositions retoquées étaient particulièrement utiles et représentaient de véritables enjeux pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs et, à travers eux, pour l'ensemble du monde agricole et rural. rural. Que fallait-il faire alors ? L'ensemble de ces dispositions ne pouvant être rassemblé dans une thématique suffisamment réduite pour constituer une proposition de loi homogène, j'ai souhaité constituer, parmi les articles retoqués de la loi Égalim, la loi Égalim, un ensemble d'articles cohérents et efficaces, visant à la fois à protéger le consommateur, à soutenir les producteurs et à valoriser les territoires. Il m'est alors rapidement apparu que se focaliser sur les dispositions en lien avec les signes et mentions valorisantes permettait de répondre à l'ensemble de ces objectifs. Sur cette base, j'ai proposé une ébauche de texte à plusieurs de mes collègues, que j'ai souhaité associer à l'écriture de cette proposition de loi, à savoir Henri Cabanel, Franck Montaugé et Jean-Claude Tissot. C'est donc le résultat de ce travail collectif que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Afin de ne pas dénaturer ce texte et, surtout, de permettre sa transmission à l'Assemblée nationale, nous avons fait le choix de le limiter à quatre dispositions qui concernent plusieurs filières agricoles- miel, fromage, vin -et touchent tous les territoires. Seul l'article 2 peut être considéré comme plus spécifique, puisqu'il concerne la Clairette de Die, production emblématique du département de la Drôme dont je suis élue. Il répond aussi à une demande des producteurs en faveur d'une adaptation des signes valorisant cette production aux nouveaux enjeux du XXI siècle. J'ai accepté que mon collègue sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet puisse joindre l'examen de sa proposition de loi sur la Clairette de Die à celui de la nôtre, car son texte est identique à l'article 2, et il aurait été dommage que nous ne nous retrouvions pas sur ces enjeux qui dépassent les clivages politiques. D'ailleurs, je ne doute pas que notre autre collègue sénateur de la Drôme, Bernard Buis, élu dans le Diois, apportera aussi son soutien. Au-delà de cet article, mes chers collègues, l'ensemble des dispositions que nous proposons vous sera présenté dans le détail par les rapporteurs Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel, dont je salue le précieux travail réalisé dans un esprit constructif, qui a permis d'affiner la rédaction du texte. Le monde change, les préoccupations de nos concitoyens. Ainsi, les modes de consommation évoluent. Nous assistons depuis plusieurs années non seulement à la montée en puissance d'une exigence de traçabilité, de transparence et de qualité des produits, mais aussi à une attente forte des consommateurs d'une information juste et claire sur les produits alimentaires qui sont consommés au quotidien et sur les conditions de leur production. Ce sont au moins huit consommateurs sur dix qui souhaitent plus de transparence pour les produits alimentaires et près de 80 % des personnes qui se déclarent prêtes à payer plus cher pour un produit régional ou pour un produit 100 % français. Cette exigence accrue d'éthique dans l'alimentation est tout particulièrement ressortie au cours des États généraux de l'alimentation et, bien entendu, des débats de la loi Égalim. Les mentions et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits sont parmi les moyens les plus efficaces pour répondre à la fois aux demandes de transparence et de traçabilité et à la à la recherche de saveur et d'authenticité des productions. Toutes les dispositions que nous avons reprises dans cette proposition de loi, que ce soit les informations figurant sur les étiquettes- miel, vin -ou l'adaptation de certaines mentions valorisantes- fromage fermier, appellation Clairette de Die -contribueront à restaurer durablement une relation de confiance entre les producteurs et les consommateurs. L'agriculture française est confrontée à une concurrence internationale, parfois déloyale, face à laquelle il est nécessaire de promouvoir les signes et mentions valorisantes. Les producteurs français sont désireux de faire reconnaître, protéger et valoriser la qualité de leur production, leur savoir-faire et leurs territoires. Ainsi, il convient de mieux mettre en valeur les garanties de leurs produits en termes d'origine et de qualité, grâce aux signes et mentions valorisantes, qui contribuent, en outre, à permettre une meilleure rémunération et une meilleure reconnaissance de leur travail. Certaines dispositions de notre texte soutiennent donc les productions sous signe et indication de la qualité et de l'origine, ou qui garantissent l'origine géographique ou les modes de production. Les SIQO ont l'avantage d'être facilement reconnus par les consommateurs, qui, s'ils ignorent parfois leurs caractéristiques et leurs garanties exactes, savent que ces mentions constituent une certaine assurance-qualité des produits sur lesquels elles sont apposées. L'étiquetage des produits alimentaires, plus généralement l'information sur les produits, permet de faire évoluer les pratiques. Le pari est que, avec davantage d'informations en leur possession, les consommateurs feront des choix plus éclairés et privilégieront l'agriculture française, notamment l'agriculture paysanne. en effet, à travers cette proposition de loi, il s'agit toujours de soutenir le modèle agricole français qui, à côté des grandes cultures, développe une agriculture de terroirs, basée sur le savoir-faire de nos producteurs et la valeur ajoutée de nos produits. Ce modèle offre des garanties de qualité incontestables. Les filières agricoles et alimentaires concernées par ce texte sont parmi celles qui contribuent au dynamisme de nos territoires ruraux et à leur attractivité économique et touristique. Les consommateurs français mais aussi étrangers plébiscitent les produits clairement identifiés. À travers les mentions et signes de la qualité et de l'origine, ce ne sont pas seulement les produits agricoles ou alimentaires français qui sont valorisés, mais aussi les territoires où ils sont produits et toute l'économie rurale qu'ils contribuent à entretenir. Mettre en valeur les productions locales, les circuits courts, la territorialisation de l'alimentation constitue un puissant puissant levier permettant de soutenir l'économie locale, mais aussi de préserver notre environnement et de tendre vers la nécessaire transition agroécologique. C'est là une demande de nos concitoyens et des consommateurs en général, mais c'est aussi une orientation générale plus que souhaitable de notre agriculture et de notre société. Au fond, c'est un trio gagnant que doivent former les consommateurs, les professionnels et les territoires. J'espère que le Sénat saura parvenir à un consensus un consensus et que ces mesures de bon sens trouveront une issue favorable, pour une mise en application la plus rapide possible. La parole

Le Conseil constitutionnel a confirmé, d'un point de vue juridique, que la plupart des articles ajoutés à la loi Égalim n'avaient pas de lien, même indirect, avec le format initial du projet de loi. Il a censuré près d'un quart Certains articles censurés avaient toutefois fait l'objet d'un travail approfondi et consensuel entre nos deux assemblées et répondaient à des attentes tout à fait légitimes et justifiées de nos territoires. Les deux propositions de loi que nous examinons, celle de Marie-Pierre Monier et celle de Gilbert Bouchet, dont je salue le travail, ont justement pour objet de reprendre ces principales dispositions sur l'étiquetage et les mentions valorisantes. La proposition de loi de Marie-Pierre Monier entend permettre l'étiquetage de certains fromages fermiers affinés en dehors de la ferme et renforce l'information du consommateur sur l'origine des produits qu'il achète, notamment les pots de miel et les bouteilles de vin. Enfin, tout comme la proposition de loi de Gilbert Bouchet qui a, en conséquence, été intégrée à ce texte, elle permet aux producteurs du Diois de diversifier leur production.

depuis un arrêt du Conseil d'État de 2015, il n'est plus possible pour les producteurs de fromages fermiers ne disposant pas de cave d'affinage au sein de leur exploitation de mentionner que leurs fromages sont fermiers. Cet arrêt met en péril de nombreuses petites structures de nos territoires en empêchant les producteurs de valoriser au mieux leurs produits. Certes, il faut protéger la mention valorisante « fromage fermier »- de cette proposition de loi -, afin qu'elle ne soit pas dévoyée, mais ce n'est pas en écartant certains producteurs plutôt que d'autres, notamment les producteurs qui répondent aux critères de production des fromages fermiers, que nous y parviendrons. La commission proposera de revenir à la rédaction issue de la loi Égalim en ajoutant une sécurité supplémentaire, suggérée par notre collègue Pierre Louault, la mention du nom du producteur sur l'étiquette, afin de s'assurer que la production demeure bien sous la responsabilité directe du fermier. Enfin, les miels donneront probablement lieu à un débat important. Il est anormal que le consommateur ne puisse pas connaître l'origine des miels qu'il achète. La directive européenne offre déjà la possibilité d'afficher tous les pays d'origine, mais elle n'est malheureusement pas ou peu appliquée en France. C'est pourquoi nous proposons de l'inscrire explicitement dans la loi. Juridiquement, il est difficile d'aller plus loin, sauf à négocier à l'échelon européen un renforcement de la fiabilité des étiquetages des miels. Nous savons que ce point est très attendu des consommateurs. Aussi, monsieur le ministre, afin de vous aider dans cette négociation qui, nous le savons, vous tient à coeur, la commission proposera une solution opérationnelle

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues,

vous rappellera quelques souvenirs sur ces bancs. Anne-Catherine Loisier a rappelé les principaux éléments relatifs à l'étiquetage du miel et des fromages fermiers. Passons aux problématiques viticoles auxquelles les deux propositions de loi entendent répondre. L'article 2 entend abroger une L'article 2 entend abroger une vieille loi de 1957, qui interdit aux producteurs de l'AOC Clairette de Die de produire d'autres vins mousseux. Il est en tout point identique à l'article que nous avions adopté lors de la loi Égalim. Depuis une douzaine d'années, force est de constater que la couleur rose a le vent en poupe Je veux bien sûr parler des vins, qu'il s'agisse des vins tranquilles ou des effervescents ! La France est le premier producteur mondial de rosé, avec une augmentation de ses volumes de 50 % en dix ans. Pourquoi les producteurs de l'Est pourraient-ils faire du vin mousseux blanc ou rosé selon leur choix et non les producteurs de la zone de Die ? L'article 2 permettra aux producteurs du Diois pourront le faire. En revanche, ils ne pourront produire que du vin mousseux rosé sans appellation.

Une vaste tromperie a été décelée en grande surface, surtout pour les de vin d'une contenance de deux à dix litres. Le consommateur est leurré avec des imageries régionales, un nom francisé, un cépage, mettant en avant le conditionnement français, alors que ces vins sont étrangers, notamment espagnols.

les services des fraudes pour leur demander des contrôles accrus. Le procédé est une astuce de contournement du droit européen : l'obligation d'informer sur le pays d'origine est bien respectée. Elle figure bien avec toutes les autres mentions obligatoires, dans la police exigée par la réglementation européenne. Reste que cette information se retrouve le plus souvent dissimulée sur la face cachée du, donc non visible par le consommateur. Dans un autre registre, que vaut la mention France avec une taille de caractère de 1,2 millimètre, la grande image d'un paysage provençal sur toutes les faces ? Il est urgent d'agir. La réglementation en vigueur prévoit déjà tous les instruments pour lutter contre ces méthodes. L'enjeu est donc non le droit, mais la pratique : la pratique commerciale trompeuse est déjà contrôlée par la DGCCRF et peut donner lieu à des sanctions pénales, mais ces contrôles ne sont pas assez nombreux pour endiguer ce phénomène. la commission, plusieurs responsables professionnels m'ont indiqué le manque de moyens de ces services : moins d'une dizaine d'agents, m'ont-ils dit, pour le territoire de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Monsieur le ministre, la filière est unanime pour travailler dans le sens d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement et engagée dans des signes de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs. Cependant, comment soutenir cette volonté s'il n'y a pas suffisamment d'agents pour contrôler et dissuader les distributeurs peu scrupuleux ?

Le fait de clarifier l'article 4 rassurerait les producteurs et irait dans le sens que nous souhaitons tous, à savoir une meilleure transparence pour le consommateur. À l'échelon international, la France conserve encore l'image du Pays des Vins de qualité, car nous avons créé l'appellation d'origine contrôlée et l'indication géographique protégée. Dans les deux cas, les mots « contrôlée » et « protégée » sont les garants d'une qualité et d'une sécurité fortes. Monsieur le ministre, quels moyens allez-vous développer et déployer pour garantir cette excellente image de la France ? La

pas suffisant. Espérons que, dans les mois et les années qui viennent, la situation s'améliore. Les ordonnances qui ont été prises sur le seuil de revente à perte, sur les prix anormalement bas,

Je n'en suis pas totalement sûr, et la démonstration doit en être faite. Je pense au contraire que nombre de nos concitoyens n'ont absolument pas les moyens de payer plus cher leur alimentation.

J'ai coutume de rappeler que ce que nous trouvons sur les rayons des grandes surfaces ou dans nos marchés, ce n'est pas ce que cela coûte, mais c'est ce que cela vaut.

que je n'ai jamais opposées entre elles : l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, les circuits lents et les circuits courts, l'agriculture productive et l'agriculture des marchés paysans. Nous avons besoin de toutes ces agricultures. C'est ainsi que nous y arriverons.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Gremillet. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues,

Si je les évoque en cet instant, c'est parce qu'il nous faut retrouver une certaine forme d'honnêteté, mais surtout d'efficacité.

simple : l'ensemble des produits qui seront vendus en Europe et en France doivent correspondre aux exigences que nous leur imposons. La

madame la présidente de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un texte reprenant quatre articles de la loi Égalim, lesquels avaient fait, à l'époque, l'objet d'un certain consensus, et je m'en réjouis. Fruit d'un travail parlementaire fourni et de longs mois de débats, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

À mon sens, il aurait fallu étendre davantage le champ de cette proposition de loi et y inclure d'autres mesures qualifiées de « cavaliers » par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi, et je tiens à le souligner ici, un groupe de travail parlementaire de La République En Marche, auquel j'appartiens, a également travaillé sur un texte portant la même ambition. Il a été déposé à l'Assemblée nationale le 20 mars dernier. Mes chers collègues, les États généraux de l'alimentation et les trois mois de concertation et d'échanges ont permis d'aboutir à un constat nécessaire de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs en termes de qualité des produits ou de respect de l'environnement. Les mesures visant à améliorer la transparence sur les conditions et les lieux de production de nos produits agricoles ont ainsi une double ambition : protéger le consommateur en lui offrant une meilleure information sur ce qu'il mange, mais aussi- dois-je le rappeler ? -protéger nos agriculteurs. Tous les signes et mentions de la qualité et de l'origine jouent en faveur de notre production nationale. Les produits de nos terroirs sont une garantie d'excellence pour le consommateur. Une meilleure information valorise nos produits et fait ainsi gagner des parts de marché à nos agriculteurs. Venons-en au fond du sujet. sujet. L'article 1 de la proposition de loi porte sur la labellisation des fromages dits « fermiers », la situation actuelle n'étant pas acceptable. Les fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage. Or, nous le savons, les affineurs ont historiquement été à l'origine de la création de nombreuses appellations d'origine contrôlée. Dès lors que le lien direct du producteur avec le produit final et la mise en oeuvre de pratiques traditionnelles d'affinage

cela reviendrait à exclure les petits producteurs, qui peinent à valoriser leurs produits. Le dispositif proposé permettrait de mettre fin à l'insécurité juridique. porte sur l'étiquetage de la mention du pays d'origine des mélanges de miels issus de plus d'un pays, était attendu de longue date par nos producteurs, qui subissent la concurrence européenne et internationale. En 2017, quelque 20 000 tonnes de miel ont été produites en France et 35 000 tonnes ont été importées, mais aucune indication du pays d'origine n'apparaît sur les étiquettes.

Toujours dans un souci de transparence et de bonne information des consommateurs, mais aussi afin de mettre en valeur nos productions françaises, nous nous devons d'être plus ambitieux C'est pourquoi nous sommes favorables à l'inscription par ordre décroissant des pays d'origine. Cette négociation doit également être portée à l'échelon européen afin de soutenir une filière en grande difficulté, confrontée au déclin du nombre d'abeilles dans l'Hexagone. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous.

Si l'on considère que le droit en vigueur est suffisant, les contrôles sont, quant à eux, largement déficients. Les étiquettes de certains vins issus de pays étrangers donnent à penser qu'ils ont été produits en France à partir de récoltes du vignoble français. C'est de la fraude, oui, et le consommateur est trop fréquemment induit en erreur Ces pratiques sont préjudiciables à toute une filière, laquelle est importante, puisqu'elle représente 15 % de la production agricole française. La clarification des règles d'étiquetage et l'indication visible de la provenance de ces vins sont donc primordiales pour assurer l'information claire et loyale du consommateur. Nous vous interpellons aujourd'hui, monsieur le ministre, sur le manque de moyens alloués aux contrôles de la DGCCRF, Enfin, mes chers collègues, je regrette que les amendements sur le maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte viticole, très largement soutenus, aient été déclarés irrecevables par la commission des affaires économiques. je suis heureuse que le sujet ait été repris par nos collègues députés à l'article 8 de leur proposition de loi. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour vos propos. En effet, les agriculteurs, notamment les éleveurs, doivent décider du prix de vente de leurs produits, et non pas le subir.

par le Conseil constitutionnel. Cette proposition de loi a donc plusieurs objectifs : il s'agit de permettre une certaine diversification des productions, une valorisation de certains signes de qualité et une information plus éclairée des consommateurs. Dans les faits, il s'agit de continuer à protéger certaines appellations d'origine, tout en permettant aux agriculteurs de valoriser des productions qui ne correspondent pas forcément aux cahiers des charges.

L'article 2 abroge la loi de 1957, qui interdisait aux viticulteurs de produire d'autres vins mousseux que de la Clairette de Die au sein de l'AOC du même nom.

l'indication obligatoire du pays d'origine des vins, afin de permettre une information éclairée du consommateur et de lutter contre les contrefaçons indications abusives d'origines. Si nous partageons l'objectif central de ce texte, nous devons cependant veiller à ce qu'il ne dénature pas la protection accordée à certains produits ; je pense au label fermier pour les fromages.

d'une extension du label « fromage fermier » aux fromages ne bénéficiant pas d'un signe de qualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre groupe n'avait pas voté l'article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, laquelle renvoyait à « la notion d'usages traditionnels

Ils favorisent la variété et la diversification de la production. Ils protègent bien évidemment les bassins de production traditionnels, valorisent le savoir-faire des agriculteurs, et permettent aux producteurs de commercialiser des produits différenciés ayant des caractéristiques clairement identifiables.

Ainsi, le Canada n'a reconnu que des indications protégées européennes. Sur près de 1 400 IGP, seuls 173 produits ont été reconnus. En outre, la protection qui leur sera accordée est loin d'être absolue, puisque le Canada a négocié le maintien provisoire ou définitif

le sujet abordé dans cette proposition de loi est essentiel. La bonne information du consommateur est nécessaire, à la fois pour répondre à une demande légitime de transparence sur l'origine et la fabrication des produits, mais aussi parce qu'il s'agit d'un réel levier pour changer les modes de production et évoluer vers des pratiques plus vertueuses. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter, par leur acte d'achat, valoriser les producteurs qui s'engagent pour la qualité et pour le respect de l'environnement et de la biodiversité, les deux étant très liés.

comme cela a déjà été indiqué, le Conseil constitutionnel a estimé que ces articles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte. J'ai été, pour ma part, sidéré- il n'y a pas d'autre mot -par cette décision. Comme je l'ai dit, la bonne information du consommateur et les mentions valorisantes sont des leviers indispensables de la transition de notre agriculture.

C'est d'autant plus nécessaire que certaines mesures me paraissent urgentes, notamment l'étiquetage de l'origine des miels. En effet, nous connaissons tous les difficultés de nos apiculteurs, affectés par les fortes

des miels qu'elle consomme. Et, nous le savons, certains pays pratiquant des prix extrêmement bas sont trop souvent épinglés pour des fraudes, comme l'ajout de sirop de sucre. Dans ce contexte, le consommateur ne dispose même pas de l'information minimale, la pratique des mélanges de miels permettant jusqu'à présent d'échapper à l'obligation de mentionner l'origine du produit. Pour ma part, je trouve que le mélange de miels d'importation devrait être remis en cause

on nous a opposé le droit européen, qui nous empêcherait d'adopter l'affichage du pourcentage. Or il est déjà pratiqué par la Grèce depuis 2011 et les Espagnols se préparent à l'adopter Par ailleurs, je suis convaincu que voter cette mesure aujourd'hui ne pourra que contribuer à accélérer un changement à l'échelon européen. La France doit être leader pour faire bouger l'Europe, parce que l'Europe doit bouger.

cela ne vous surprendra pas de ma part, à l'étiquetage des huîtres, selon qu'elles soient nées en mer ou en écloserie. Ce sujet n'a pas été repris dans la proposition de loi, et je le regrette.

Je proposerai également un amendement visant à aller plus loin s'agissant de la protection de la mention « fromage fermier. » En effet, cette mention doit pour moi rester attachée, comme c'est le cas aujourd'hui, aux fromages affinés à la ferme. Il s'agit d'éviter une banalisation de cette mention valorisante. En nous appuyant sur la position des producteurs de fromages fermiers, nous proposerons qu'elle soit autorisée pour l'affinage à l'extérieur de la ferme seulement pour les mentions liées à l'origine, qui garantissent un véritable lien au terroir, et à condition que le nom du producteur soit indiqué sur l'étiquette. La rédaction actuelle pourrait entraîner des dérives. On sait déjà que l'industrie, dont Lactalis, a racheté des structures d'affinage, afin de récupérer cette mention valorisante. Pour finir, cette proposition de loi, qui vise à renforcer l'information du consommateur, va dans le bon sens : promouvoir, l'information du consommateur, la qualité et le lien au terroir est est vertueux. Toutefois, un risque d'appropriation par l'industrie pèse sur ces mentions valorisantes. Comme pour l'agriculture biologique, il faut défendre une forte exigence des mentions valorisantes, sous peine de pénaliser l'ensemble des filières.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, l'agriculture française est riche de ses nombreux producteurs. Dans toutes les régions, ceux-ci sont passionnés par leur métier, produisant des produits de qualité reconnus dans le monde entier. L'excellence alimentaire française est renforcée par les signes et les labels de qualité. Ces emblèmes de notre modèle connaissent un succès croissant, en réponse à une demande accrue de qualité de la part des consommateurs. D'après un recensement agricole récent, 49 000 exploitations agricoles réalisent au moins une production sous AOP, IGP ou label rouge, hors produits viticoles. S'y ajoutent 76 500 exploitations viticoles et plus de 25 000 exploitations engagées en agriculture biologique. Au total, près de 30 % des exploitations françaises sont concernées par les signes d'identification de la qualité et de l'origine, ou SIQO. C'est considérable, et ce doit être un motif de fierté nationale. Nous devons les encourager, les soutenir, les promouvoir Ces labels français et européens présentent en effet de nombreux avantages : d'une part, la garantie de la qualité, de la provenance et des méthodes de fabrication pour le consommateur ; d'autre part, une meilleure visibilité, une reconnaissance d'un travail de qualité, ainsi qu'une meilleure rémunération pour le producteur. Il faut, en contrepartie, veiller à la pertinence de ces labels et signes de qualité, adaptés pour ne pas induire en erreur le consommateur. C'est le sujet de l'article 1, visant à préciser l'emploi du label fermier. Je soutiens cette démarche elle s'inscrit dans le cadre d'un dialogue ouvert et transparent avec toutes les parties intéressées et ne dénature pas le sens de ce label, assurant ainsi une bonne information du consommateur. l'adapter à la réalité du terrain tout en préservant les intérêts de ces producteurs fermiers. Présents dans tous les territoires, ils participent à la richesse de la gastronomie française. Il doit ainsi être indiqué clairement sur l'avant de l'emballage des produits à la fois le nom du producteur et celui de l'affineur. L'article 3 concernant le miel va également dans le bon sens. Réclamé par le secteur apicole, le groupe Les Indépendants - République et Territoires l'avait déjà défendu lors de la discussion du projet de loi Égalim, par la voix de ma collègue Colette Mélot. Nous défendrons les producteurs français, alors que le miel est une denrée de plus en plus convoitée par les Occidentaux. Entre 2008 et 2015, sa production mondiale a augmenté de 8 %, et les exportations de 61 %. Depuis 2015, de nombreux pays européens ont accru leurs exportations de miel, mais aussi leurs importations en provenance de Chine. En France, plus de la moitié du miel consommé sur le territoire est issu de l'importation. Cette situation peut impliquer des méthodes trompeuses. Ainsi, quelque 45 % des miels seraient d'une origine différente de celle mentionnée sur le pot, pot, sans parler des mélanges au glucose, des miels dilués à l'eau et autres mélanges de miels divers et variés. Pour contrer ces méthodes trompeuses et mieux protéger le miel, il est important de rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine des miels issus de mélanges de productions, et ce en ordre décroissant. L'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé sera ainsi connu des consommateurs. Nous protégeons donc les producteurs français, tout en valorisant un miel de qualité. Le sujet de l'étiquetage des miels est similaire à celui des vins. Lorsque nous touchons au patrimoine national, nous nous devons de réagir, tout d'abord en condamnant les actes frauduleux trompant l'État français et les consommateurs. La pratique de la naturalisation du vin espagnol, devenue courante, est ainsi inadmissible : on parle de 10 millions de bouteilles de rosé ! Les outils pour combattre ces actes délictueux existent. Les agents de la répression des fraudes contrôlent régulièrement les importateurs français de vins étrangers, mais le constat est là. Le dispositif en place est-il assez dissuasif ? Nous devons adopter de nouveaux outils législatifs. Nous devons aussi, et avant tout, renforcer l'application du dispositif existant pour combattre ces tromperies des consommateurs. Bien entendu, la priorité doit rester la bonne information du consommateur. Ce dernier doit être en mesure de faire des choix, en ayant toutes les informations nécessaires quant à la qualité et la provenance. Un contrôle plus strict de l'étiquetage serait souhaitable, notamment en mentionnant l'origine de chaque côté du contenant. L'offre gagnerait d'ailleurs en clarté si les revendeurs évitaient toute confusion dans leurs rayons en séparant clairement les vins français des vins étrangers. Ces mesures permettent donc de compléter la loi Égalim et d'envoyer un message sur l'importance de la défense des productions agricoles françaises. C'est une force de notre pays qu'il nous revient de promouvoir. C'est aussi une façon de renforcer la bonne information du consommateur, lui permettant ainsi de faire des choix alimentaires éclairés. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires est favorable à cette proposition de loi avec les amendements proposés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, chers collègues, nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à avoir regretté que la loi qui devait décliner les états généraux de l'alimentation ne soit pas allée plus loin. Finalement, la loi Égalim n'aura permis ni de garantir un revenu réellement rémunérateur pour les agriculteurs ni d'améliorer réellement l'accès à une alimentation saine, durable et de qualité. Il était donc d'autant plus regrettable que les quelques avancées obtenues au cours de nos travaux aient été retoquées par le Conseil constitutionnel, pour une raison de forme. Il n'était bien évidemment pas possible pour nous de nous pencher de nouveau sur l'ensemble des dispositions rejetées. Avec cette proposition de loi, notre collègue Marie-Pierre Monier nous invite donc à nous concentrer sur l'amélioration du dispositif relatif aux signes de qualité et d'origine. Cette démarche me semble tout à fait pertinente, les SIQO étant fortement emblématiques de ce que nous voulons pour l'agriculture et l'alimentation de demain. Ils permettent en effet de valoriser la qualité des produits, le savoir-faire de nos producteurs, y compris à travers le prix de vente. Avec les SIQO des produits fermiers, seul le producteur reçoit le bénéfice de la plus-value dont il est à l'origine. Ils constituent aussi l'une des réponses à la demande croissante des consommateurs d'une plus grande transparence en matière de qualité et de sécurité alimentaire. Plusieurs des dispositions de ce texte sont ainsi très attendues par les agriculteurs. La plupart de ces mesures avaient été adoptées à une large majorité, tant dans cette chambre qu'à l'Assemblée nationale. Elles ne devraient donc pas susciter de clivage politique profond entre nous. D'ailleurs, j'imagine que nos collègues du groupe Les Républicains, en saisissant le Conseil constitutionnel, n'avaient pas particulièrement l'intention de faire tomber ces dispositions, qu'ils avaient eux-mêmes soutenues. Le choix, inhabituel pour un texte qui ne comporte que cinq articles, de deux corapporteurs, issus l'un de notre groupe et l'autre de la majorité sénatoriale, marque cette volonté de parvenir à un consensus large sur cette proposition de loi. Henri Cabanel et Anne-Catherine Loisier, qui étaient rapporteurs de ces mêmes articles pour la loi Égalim, pourront ainsi enrichir nos débats de leur expertise. Nous aurons peut-être des divergences sur la rédaction « technique » de ces articles, notamment à l'article 4, mais nous souhaitons réellement parvenir à un accord, afin que les SIQO puissent bénéficier de la juste reconnaissance que cette proposition de loi peut leur apporter. C'est aussi pour cela que nous avons fait le choix, à l'article 1 et, initialement, à l'article 3, de nous en tenir à la rédaction de l'Assemblée nationale lors de la dernière lecture de la loi Égalim. Nous souhaitions ainsi permettre à ce texte d'être le mieux armé pour affronter les écueils de la navette parlementaire. L'article 2 ne devrait pas poser de difficulté puisqu'il est rédigé dans les mêmes termes que la proposition de loi concernant la Clairette de Die de notre collègue Gilbert Bouchet, laquelle est d'ailleurs annexée au présent texte. Avec cette proposition de loi, nous avons la possibilité de mieux reconnaître et protéger des produits français qui sont constitutifs de notre patrimoine commun. Je pense, en particulier, aux vins et aux fromages fermiers. Nous avons l'occasion de redonner de la sérénité aux consommateurs qui veulent pouvoir acheter en confiance des produits de qualité, sains et au moindre impact environnemental. La question de l'étiquetage des miels en est particulièrement symbolique. Enfin, nous avons une occasion de nous appuyer sur de bonnes pratiques existantes, en les confortant, afin de faire un pas supplémentaire vers le modèle agricole que nous avons le devoir de mettre en place pour notre planète et les générations qui vont nous succéder. Pour ces raisons, mon groupe votera ce texte. La parole

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, monsieur le ministre, de l'adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. afin d'améliorer le revenu des agriculteurs et de réduire leurs contraintes réglementaires, d'une part, et de protéger l'information et la santé des consommateurs, d'autre part. L'Assemblée nationale n'a pas retenu toutes nos remarques, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a censuré quelques articles, notamment ceux qui étaient exposés dans la proposition de loi de nos collègues Marie-Pierre Monier et Gilbert Bouchet telles que l'affichage de la provenance des vins et du miel ou la notion qualificative de fromages fermiers. Les raisons invoquées pour exclure ces articles du texte voté par les députés sont qu'ils n'auraient pas de lien avec le texte visant à une alimentation saine et durable. En revanche, le Conseil constitutionnel a validé que la fin des pics à steak ou des plateaux-repas en plastique avaient, quant à eux, bel et bien un rapport avec le texte ... Soit ! Bonne remarque ! Le Sénat a pris acte de cette décision et propose de reprendre certaines des dispositions censurées. Il le fait avec un esprit d'ouverture et de consensus, puisque cette initiative législative émane des groupes socialiste et républicain et Les Républicains, et reprend quelques-unes des dispositions introduites par des membres du groupe Union Centriste. Nous travaillons donc à l'intérêt général. Si ce texte est voté, monsieur le ministre, soyez convaincant auprès de nos collègues du Palais Bourbon afin qu'eux aussi répondent à l'intérêt général. Très bien ! Tout à fait ! Si les sénateurs réintroduisent si rapidement ces mesures, c'est que leur portée est partagée et dense. D'une part, nous souhaitons protéger nos appellations dans un monde qui tend à s'uniformiser. Les fromages sont l'une des identités de notre patrimoine culinaire français. Ils font partie des ingrédients élémentaires du repas gastronomique français reconnu par l'Unesco, vous l'avez signalé, monsieur le ministre. D'autre part, il s'agit également d'assurer la compétitivité de la Ferme France, ce qui aurait dû être l'un des objectifs de la loi Égalim. La concurrence libre et non faussée est un pilier de la construction européenne et des règles qui organisent le marché commun et le commerce international. Par les dispositions présentes et par certains amendements qui seront débattus aujourd'hui, la transparence due aux consommateurs s'améliore : les producteurs français et européens pourront mettre en valeur leurs produits et se servir de cette visibilité retrouvée pour développer leur secteur et, pourquoi pas, augmenter et rendre de la valeur ajoutée à leurs productions. Si je prends l'exemple du miel, traité à l'article 3, la France en consomme près de 40 000 tonnes par an, ce qui la place parmi les plus forts consommateurs d'Europe. Or seulement 20 000 tonnes au mieux, soit la moitié environ, sont fournies par des apiculteurs français. La valorisation de leur gamme leur donnera un souffle nouveau. Donner des précisions sur la provenance de l'origine des miels est une idée simple et bienvenue. En effet, on pouvait lire, conformément à la réglementation : « Mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne » Autant inscrire « Miel de la planète Terre », on donnerait autant d'informations à l'amateur de produits sucrés ! Citer les pays, et cela conformément au droit européen, renverse cette tendance. Voilà une sorte de « sur-transposition » des normes européennes en France que personne ne devrait contester ! Les auteurs de la proposition de loi souhaitent également que l'étiquette d'une bouteille de vin ou de tout autre contenant comporte en évidence la mention du pays d'origine afin de ne pas induire en erreur le consommateur, même si des attributs français, comme le nom, un dessin de château, perturbent la compréhension du produit. Les rapporteurs ont estimé que l'article 4 ne changerait pas la donne. En revanche dans le rapport, une phrase m'interpelle : « La La provenance doit donc être précisée selon des formules précisées à l'article 45 de ce règlement : " vin de " ou " produit de ", suivi du nom de l'État membre où les raisins sont " récoltés et transformés en vin

si l'Europe est souveraine pour l'inscription de la décroissance des ingrédients d'un bien de consommation sur une étiquette, on peut comprendre que nos concitoyens s'interrogent sur son efficacité. C'est pourquoi je maintiens que définir clairement l'origine de nos produits, notamment pour le miel, épouse parfaitement les attentes des consommateurs français et européens et ne trahit pas l'esprit de l'Union européenne de la défense du droit des consommateurs. Faire apparaître tous les pays et, de surcroît, par ordre d'importance ne choquera pas, je pense, les commissaires de Bruxelles. De plus, monsieur le ministre, je veux croire que vous serez un ambassadeur fidèle de la volonté du Parlement français de défendre les droits des consommateurs et n'aurez donc pas de mal à convaincre vos collègues européens. J'ajouterai par ailleurs que ces normes auront d'autant plus d'efficacité que les contrôles seront nombreux et coercitifs, ce qui ne manque pas d'inquiéter au regard des moyens alloués à la DGCCRF. Ce sont des mots, monsieur le ministre, que j'ai déjà prononcés lors de l'examen budgétaire, que ce soit pour le Brexit ou pour tous les autres contrôles : il faut suffisamment de vétérinaires et d'agents de répression des fraudes pour respecter les règles. Le respect des normes, c'est ce qui fait la qualité des productions et la confiance des consommateurs. Le respect des normes, c'est aussi l'expression d'un terroir et de ses produits qui peuvent être mentionnés dans le cahier des charges d'une appellation. La Clairette de Die répond à ces exigences. Un accord local semble unanime pour abroger la loi du 20 décembre 1957. S'il n'est Clairette de Die qu'en vallée de la Drôme, l'interprofession y veillera. Je n'ai que très peu de mots à dire à ce sujet puisque tout le monde semble unanime et j'imagine, monsieur le ministre, que vous avez un avis très personnel sur ce sujet. Ce menu législatif nous amène bien évidemment au fromage Les auteurs du présent texte ont voulu préciser les conditions d'usage de la mention « fermier », afin de sécuriser le cadre juridique de l'affinage extérieur à la ferme. En effet, il conviendrait de rectifier l'arrêt du Conseil d'État de 2015, qui dispose que seuls les fromages affinés sur l'exploitation peuvent bénéficier du terme « fermier », puisqu'il ne correspond pas à la réalité de certains cahiers des charges de telle ou telle appellation. Comme l'a détaillé le rapport d'Anne-Catherine Loisier, l'article 9-1 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages encadre déjà très strictement ces pratiques en réservant l'usage de la mention aux fromages fabriqués « selon des techniques traditionnelles Une loi est cependant nécessaire pour permettre de nouveau l'affichage de la mention « fromage fermier » en cas d'affinage à l'extérieur de la ferme, et les modalités techniques encadrant cet affichage sont à définir au niveau réglementaire. Monsieur le ministre, il vous appartiendra donc de prendre les dispositions administratives accomplissant la volonté du législateur. Mes chers collègues, le groupe Union Centriste se prononcera favorablement sur cette proposition de loi si celle-ci reste dans l'esprit des mesures introduites par le Sénat lors de l'examen de la loi Égalim et si les productions agricoles hexagonales sont préservées et défendues. Quelques amendements ont été déposés, dont l'adoption devrait permettre de parfaire ce texte. La parole

constitue la production principale des viticulteurs du Diois. Elle est élaborée d'après la méthode dioise ancestrale, issue de l'assemblage de muscat blanc et de la clairette blanche. En 1908, la Clairette produite était blanche ou rosée. L'appellation d'origine datant de 1910, il faut préciser que, dans le premier cahier des charges AOC de 1942, la production de rosé n'avait pas été mentionnée. En décembre 1957, date à laquelle a été votée la loi visant à interdire la production de tout vin effervescent hors AOC dans l'aire d'appellation, il est apparu nécessaire de protéger l'appellation naissante « Clairette de Die » contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « clairette muscat ». Cette proposition de loi se compose de la manière suivante : le premier article dispose que toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée Clairette de Die et « Crémant de Die » est interdite dans l'aire géographique de production concernée. L'article 3 prévoit des sanctions en cas de méconnaissance de cette interdiction. Force est de constater que, depuis cette époque, les goûts des consommateurs ont changé. Il est donc apparu normal, aujourd'hui, de permettre aux producteurs du Diois d'adapter leur gamme à la demande de la clientèle, afin de sauver leurs entreprises et de répondre aux nouveaux enjeux du XXI siècle. Ils ont souhaité produire des vins mousseux « rosés » sous appellation « AOC Clairette de Die », conscients de la nécessité d'une modification du cahier des charges de l'AOC. En 2016, cette dernière a été homologuée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et la production de ces vins effervescents rosés a donc a donc démarré. Depuis lors, deux décisions juridiques sont venues stopper ce processus. La première est celle du Conseil d'État, qui a annulé l'arrêté homologuant le cahier des charges de la Clairette de Die, mettant en graves difficultés trois cents vignerons drômois. Il leur a été demandé de cesser La seconde est intervenue à la fin de l'année 2018, à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi Égalim. Elle a entraîné la censure de l'amendement d'abrogation de la loi de décembre 1957, pourtant voté en termes identiques par les deux assemblées, au motif qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire. Face à la concurrence de pays voisins, producteurs en grande quantité de vins rosés, l'évolution législative est fondamentale pour maintenir la vitalité de cette partie de la Drôme. Conscient de cette situation délicate, je vous ai alerté dès le mois de janvier, monsieur le ministre, par le biais d'une question orale sur ce dossier que, en tant que Drômois, vous connaissez bien, et j'ai décidé de reprendre les modifications portées par l'amendement adopté dans la loi Égalim sous la forme d'une proposition de loi, afin d'attirer votre attention et celle de l'ensemble de mes collègues sur les conséquences économiques désastreuses pour la Drôme. Sur ce dossier, nous avons été entendus, je le crois, pour essayer de résoudre le problème. entendus par la Haute Assemblée, qui a bien voulu inscrire à l'ordre du jour, de façon conjointe avec Marie-Pierre Monier, et je l'en remercie, nos deux propositions de loi, prouvant qu'au Sénat nous travaillons dans un esprit constructif. entendus également sur le terrain puisque, en collaboration avec mon collègue Chaize, sénateur de l'Ain, nous travaillons, avec les représentants des fédérations de vins de nos régions respectives, à la rédaction d'un protocole d'accord permettant, d'un côté, d'écouler ce stock, et, de l'autre, de s'engager à ce qu'aucun vin effervescent de couleur rosé présenté comme de la « Clairette de Die » ou effervescent de son ressort ne soit élaboré à l'avenir en l'absence de bases réglementaires. Fort de tout cela, je vous demanderai de bien vouloir voter pour l'abrogation de cette loi du 20 décembre 1957 relative à la Clairette Die. je vous remercie

pour le citoyen qui en fait un enjeu de confiance, pour le consommateur qui s'y réfère dans son choix et pour le producteur qui y trouve le moyen de la différenciation et de la performance économique, la transparence, la traçabilité et les conditions de production sont aujourd'hui et plus que jamais au centre de l'acte commercial alimentaire. Ces principes figuraient en bonne place dans la loi Égalim adoptée, et nous avons trouvé pour le moins surprenantes les très nombreuses décisions de rejet par le Conseil constitutionnel des articles les traduisant. Montesquieu disait qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Certainement faut-il aussi saisir le Conseil constitutionnel d'une main tout aussi tremblante. Nous avons perdu du temps, le travail est à reprendre ... Soit ! Je tiens à remercier Marie-Pierre Monier, les rapporteurs Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel, ainsi que tous nos collègues qui se sont saisis de l'opportunité de cette proposition de loi pour remettre sur le métier l'ouvrage de la valorisation des produits agricoles et alimentaires. L'article 1, en complément de l'arrêt du Conseil d'État relatif à l'usage du mot « fermier », permet l'affinage extérieur à la ferme de produits sous SIQO si les liens entre les producteurs, le produit final et les pratiques traditionnelles d'affinage sont avérés. Le dispositif est offensif, tout en respectant le client final. Ce sera un progrès. L'article 2 prend en compte des productions de vins en AOC, en permettant leur adaptation au changement climatique et à l'attente des consommateurs. Du pragmatisme qui ne lèse personne et qui conforte les économies territoriales concernées, drômoises en l'occurrence. L'abrogation de la loi de 1957 ne provoquera pas la disparition de l'AOC « Clairette de Die » ou le changement de son cahier des charges. Elle permettra aux producteurs concernés de se diversifier dans une autre production, les vins mousseux rosés notamment, afin d'améliorer leurs revenus. Toutefois, et c'est essentiel, ce vin ne pourra pas être appelé « Clairette de Die », dans la mesure où le cahier des charges de l'AOC ne le prévoit pas. Ce sera un vin mousseux rosé, produit dans la Drôme, qui pourrait bénéficier d'une IGP ou d'une appellation spécifique dans cinq ans, dix ans ou plus. Pour protéger nos apiculteurs et informer le consommateur, il faut aller au-delà des strictes obligations européennes de 2001 concernant la provenance de l'UE ou hors de l'UE. Dans un contexte où la production de miel en France a été divisée par deux en quinze ans, la situation actuelle ne peut plus durer. Il y va de la survie de la filière française pour reprendre les mots du rapporteur Henri Cabanel ce matin en commission. Pour aller dans ce sens, l'article 3 précise l'étiquetage des miels par l'indication des pays d'origine et de la proportion des composants. Dans le même esprit de respect du consommateur, la provenance des pays d'origine sera indiquée sur les étiquettes des vins vendus sans indication géographique. La renommée des vins français, le travail de nos vignerons n'en seront que mieux reconnus. Aujourd'hui, en grandes surfaces, cela a été dit surtout pour les, les consommateurs sont dupés du fait que certains vins sont vendus comme français, en jouant sur l'étiquetage, le nom francisé, en mettant en valeur un cépage, alors qu'ils sont étrangers. Les cas de tromperie sont extrêmement nombreux, on le sait. Pour aller toujours dans le même sens, celui de la transparence et du respect du client, nous regrettons que, au titre de l'article 45, les amendements identiques portés par de nombreux groupes de notre assemblée et visant au maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte ne puissent être débattus et votés aujourd'hui par la Haute Assemblée. Pour terminer, je veux saluer le travail très constructif réalisé au sein de la commission des affaires économiques sur ce texte. Les échanges ont été nourris, sans qu'à aucun moment soit perdu l'enjeu d'aboutir positivement. Pour l'essentiel, ce texte permettra de progresser vers plus de transparence et de respect des consommateurs. Les acteurs des filières concernées s'en trouveront, à n'en pas douter, renforcés. Pour ces raisons, le groupe socialiste et républicain le votera. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le texte que nous avons à étudier aujourd'hui concerne diverses dispositions, issues de quatre articles du projet de loi Égalim censurés par le Conseil constitutionnel, au motif qu'ils n'avaient pas de lien direct avec le texte. Pour ma part, je concentrerai mon intervention sur l'article 2 portant sur l'abrogation de la loi de 1957 protégeant l'appellation « Clairette de Die ». En effet, cet article avait été adopté conforme par les deux assemblées. Selon les auteurs de l'amendement à l'Assemblée nationale, cette loi était certes nécessaire à l'époque pour protéger l'appellation naissante Clairette de Die contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « Clairette muscat », elle n'avait plus lieu d'être dès lors que cette protection est assurée par d'autres textes, nationaux et européens. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que ce sujet m'intéresse particulièrement, par rapport à la Clairette de Die, vin pétillant produit par les viticulteurs du Diois dans la Drôme, mais aussi et surtout par rapport à la situation conflictuelle avec les vins du Bugey notamment le Bugey Cerdon, vin mousseux rosé produit dans l'Ain, ces vins bénéficiant tous deux d'une appellation d'origine contrôlée. Nous avons eu en effet à nous opposer, sur ses bancs, pour défendre nos territoires respectifs, et pour cause Je ne reviendrai pas sur les décisions juridiques qui ont définitivement tranché les procédures engagées. Je souhaite en revanche exprimer la bonne volonté des viticulteurs, qu'ils soient de la Drôme ou de l'Ain, pour trouver des solutions communes et intelligentes à la sortie du conflit les opposant. C'est en ce sens que nous avons oeuvré, avec mon collègue Gilbert Bouchet, que je tiens ici à saluer au regard des actions que nous avons menées. Mes chers collègues, je dois néanmoins vous avouer que l'inscription de ce texte dans cette période de négociations n'a pas facilité nos discussions. Aussi, je tiens à annoncer aujourd'hui qu'un protocole d'accord a été conclu entre le Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois et le Syndicat des vins du Bugey. Il doit faire l'objet d'une signature dans les prochains jours, pour venir clore définitivement cette situation, en redonnant à chacun une stabilité et une sérénité utiles.

Je suis heureux de constater que le bon sens et le pragmatisme ont primé pour venir à bout de ce dossier important pour nos territoires. Ils mettent en valeur notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. La parole

aucun accord international, quel qu'il soit, madame Cukierman, ne remet en cause les standards européens, notamment dans l'agriculture. Il n'y aura pas de poulet aux hormones, d'antibiotiques ou quoi que ce soit d'autre. C'est absolument faux

cet article 1 vise à sécuriser le cadre juridique de l'affinage des fromages fermiers en dehors de la ferme, en comblant un vide juridique datant du 1 septembre 2015. Nous savons qu'il va susciter des débats, comme il l'avait fait lors de la loi Égalim, et que des positions différentes vont s'affronter.

à tous les fromages. D'autres, à l'inverse, trouvent cette rédaction trop laxiste et considèrent qu'elle revient à dénaturer l'appellation « fromage fermier ». Cette différence de perception se retrouve également au sein de la profession, qui apparaît relativement divisée sur le sujet. Ainsi, l'Association nationale des producteurs laitiers fermiers est opposée au fait d'ouvrir à tous les fromages fermiers la possibilité d'être affinés en dehors de la ferme. Elle nous a notamment fait part d'un phénomène actuel de rachat de petites structures d'affinage par de grands opérateurs industriels et des risques que cela représente pour la préservation de l'appellation. C'est pourquoi elle milite pour une rédaction plus restreinte de l'article 1, qui limiterait aux seuls fromages AOP ou IGP, et non plus à tous les la possibilité d'être fermiers, avec de plus la précision du nom du producteur. De son côté, le Conseil national des appellations d'origine laitières nous a transmis son souhait de ne réserver cette possibilité qu'aux fromages sous SIQO, dans une rédaction très proche de notre article actuel.

Concernant le fait d'apposer sur chaque fromage le nom du producteur, nous y étions initialement favorables. Mais après des échanges avec des producteurs et des représentants de certaines appellations protégées, comme le Picodon, nous avons convenu que cette contrainte serait difficilement surmontable pour de petits affineurs. Nous pouvons donc constater que les positions sont très partagées sur le sujet et qu'aucune solution ne satisfera tout le monde. C'est pourquoi le groupe socialiste a fait le choix de préserver cet article dans sa rédaction actuelle, dans une version que nous pourrions finalement qualifier de compromis. Il s'agit de préserver l'appellation « fromages fermiers » dans toute sa spécificité, avec un gage de qualité lié aux SIQO, tout en garantissant aux consommateurs une véritable transparence sur les produits qu'ils consomment. En effet, soyons très vigilants à ne pas dévoyer le sens de l'appellation « fromage fermier ». Si un consommateur venait à se rendre compte que le fromage qu'il achète fermier est affiné, d'une part en dehors de la ferme, et, d'autre part, par de grands groupes industriels, c'est toute l'appellation qui pourrait en souffrir. Les mots ont un sens, et nous ne pouvons pas faire comme si les consommateurs étaient hermétiques à cette question.

d'illusionniste. En effet, que le prix soit construit dans un sens ou dans l'autre, les cours et les méthodes de la grande distribution restent les mêmes. Croire

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

ce qui pose plusieurs problèmes pratiques. Tout d'abord, cela revient à privilégier certains producteurs au détriment d'autres. Pourquoi privilégier ainsi les producteurs bio, dont le cahier des charges est bien moins précis que celui des AOP, et non les petits producteurs affiliés à de petites coopératives de nos territoires, qui produisent du fromage non AOP ? Pourquoi exclure les petits producteurs, qui n'ont pas de cave d'affinage chez eux, de la seule possibilité de valoriser leurs produits dont ils disposent ? La rédaction retenue peut même se retourner contre les producteurs sous AOP et aboutir à des cas difficilement justifiables. Imaginons par exemple un producteur sous AOP qui, une année, dépasserait légèrement les quotas. Les mêmes fromages, absolument identiques, seraient étiquetés différemment, les uns sous AOP « fermier », les autres

pour s'assurer que le fromage fermier reste sous la responsabilité du producteur lorsqu'il est affiné à l'extérieur de la ferme. L'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de la ferme devra préciser à la fois le nom de l'affineur, comme c'était le cas avant avant l'arrêté de 2015, mais également le nom du producteur. Je précise que l'affineur doit déjà lier, au nom de la traçabilité, les fromages à leurs producteurs. Le coût supplémentaire sera donc limité.

été enrayée par la mise sur le marché, en 2018, de la Clairette rosée, qui est aujourd'hui interdite. Le salut des viticulteurs du Diois passe par la possibilité de produire et de commercialiser ce vin effervescent rosé au plus vite.

Il faut rapidement abroger cette loi et donner la possibilité aux viticulteurs du Diois de produire un vin effervescent rosé qui, même s'il ne s'appelle pas Clairette rosée, permettra sans doute d'offrir une nouvelle lisibilité et un espoir pour ce territoire et ses habitants. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent,

Autrement dit, on produit quelque chose dans l'illégalité la plus totale, et, quelques années après, on fait changer la loi, entre le miel et le fromage ... Il est dommage, monsieur le ministre, que vous ne soyez pas originaire de l'Ain ! Je pense que vous m'auriez mieux comprise.

en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable. Aujourd'hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables »- le lait, les fruits ... -et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés par la loi. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut se révéler trompeuse pour le consommateur. Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio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

La réglementation espagnole irait même plus loin, en imposant que soient clairement indiqués sur l'étiquette le pourcentage de chaque miel et sa provenance- d'ailleurs, j'ai

qu'il est impossible d'aller plus loin que cet affichage de tous les pays d'origine. Toutefois, comme cela a été évoqué, un certain nombre de pays, notamment l'Espagne, se sont engagés dans une modification de leur réglementation, qui n'est pas aujourd'hui validée au niveau européen, les négociations étant en cours.

Monsieur le ministre, il semble que vous vous soyez engagé devant l'Assemblée nationale à aller plus loin, en vous déclarant favorable à un affichage plus précis et plus strict des mélanges de miels. Dès lors, la commission saisit la balle au bond et propose de graver dans la loi, avec cet amendement, l'engagement d'un affichage par ordre décroissant. Il s'agit d'un mandat minimal, nous en sommes bien conscients, que vous donnent les territoires et nos concitoyens pour améliorer l'étiquetage de nos miels.

nous soyons obligés de nous mettre au garde-à-vous devant les directives européennes. À un moment donné, il faut faire bouger les choses et nous ne serons pas les premiers, car d'autres pays européens ont déjà montré l'exemple. À nous de les rejoindre pour tirer l'Europe vers le haut.

nous prémunir contre les fraudeurs et les produits falsifiés. Certains introduisent des sucres venant d'autres types de productions et il convient de repréciser comment se détermine un miel et quelle est sa composition.

ont cherché à respecter cet équilibre entre les règles communautaires et les possibilités d'adaptation du droit en fonction du principe de subsidiarité. La définition que je vous propose d'adopter est bien évidemment conforme, car elle n'est que l'expression directe de l'annexe I, point 1, de la directive 2014/63/UE. Excusez ces précisions ... Je peux la mettre à la disposition de celles et ceux qui voudraient la comparer à la définition de mon amendement. Elles sont semblables ! Il s'agit donc de donner force de loi à cette définition. En effet, un simple décret de 2003 reprend la définition de la directive qui correspond à celle que je vous propose.

définit le miel, ainsi que ses caractéristiques de composition, dont la teneur en sucre. Cette définition est plus précise que celle qui est proposée par votre amendement. Telles sont les raisons pour lesquelles je partage l'avis de

de vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, je vais voter cet amendement.

cela veut dire que lorsque le décret et les normes seront définis au niveau européen, le ministre devra revenir devant le Parlement pour rectifier la loi. Une

Mme Dominique Estrosi Sassone. Le miel, encore et toujours ! Cet amendement vise à appuyer une recommandation de la DGCCRF relative à la dénomination de vente du miel qui qui peut préciser une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale, ainsi qu'à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. De plus, cette mention serait facultative pour ne pas alourdir les obligations des producteurs, mais sans être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les qualités du produit. Un décret du ministère de l'agriculture fixerait ainsi les critères spécifiques de qualité, d'identification et d'origine de miel qui peuvent donner droit au label. Cet amendement vise donc bien à protéger les producteurs français et à mieux lutter contre les miels d'assemblage ou ceux dont la traçabilité est impossible. Il n'est pas question de bloquer la vente de miel étranger sur le marché français, mais bien de donner plus de garanties aux producteurs français et de possibilités pour mettre en avant leur travail et assurer une transparence optimale sur des produits proposés à la vente. est l'avis de la commission ? Il s'agit de préciser des mentions facultatives sur l'étiquetage du miel, sachant que les deux points soulignés sont déjà satisfaits par le droit existant. Néanmoins, la commission a émis un avis favorable.

parcourus par son alimentation entre le lieu de production de la matière première et le lieu de transformation, jusqu'à son lieu de consommation. Enfin, pour des raisons sanitaires et afin de garantir la bonne traçabilité de ces produits,

sur les importations

proposer un compromis à nos collègues qui demandent la suppression de cet article. Je vous le précise d'emblée, l'amendement que nous avons déposé sur cet article a reçu l'accord de la que nous vous proposerons traduit toujours l'objectif de la proposition de loi, à savoir la lutte contre les pratiques trompeuses visant à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du vin. L'article L. 413-8 du code de la consommation, que nous proposons de modifier, dispose en effet qu'il est interdit de laisser penser qu'un produit a une origine française alors que tel n'est pas le cas. Une dérogation est toutefois prévue si le pays d'origine figure sur l'étiquette de manière apparente.

face à une tentative de tromperie du consommateur. Cette situation est encore plus critique lorsqu'il s'agit de. Nous avons parfaitement conscience, monsieur le ministre, que la meilleure des réponses serait un renforcement des moyens dont dispose la DGCCRF pour lutter contre les fraudes.

sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit. Si chacun s'accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires. Je considère que notre arsenal législatif et réglementaire offre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre des pratiques trompeuses en matière d'étiquetage de l'origine. Monsieur le ministre, comme Roland Courteau vient de le rappeler, il convient surtout de veiller à ce que les services de l'État en charge des contrôles disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions, particulièrement lorsque celles-ci ont été élargies du fait de l'adoption de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. tous. Si l'intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d'information des consommateurs est fort louable, nous devons veiller à ne pas surcharger notre droit de diverses dispositions, en contradiction, par ailleurs, avec notre objectif permanent de simplification. Tel est l'objet du présent amendement.

un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Cette interdiction de tromper le consommateur est donc déjà prévue noir sur blanc. Toutefois, l'alinéa suivant précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents,

pour des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale. Il est question, notamment, de l'emploi des termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale. En effet, de telles dénominations entretiennent la confusion dans l'esprit du consommateur, voire introduisent un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens. Je vous propose donc d'intégrer à ce texte un article qui participe de la bonne information du consommateur sur l'origine, animale ou végétale, des produits qu'il consomme. Quel est

L'utilisation du glyphosate dans l'agriculture française est source de controverses depuis plusieurs années. La stratégie de la France pour sortir de cet herbicide ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs, qui n'auraient pas de produits de substitution et subiraient des distorsions de concurrence avec les autres pays européens. Le 7 mars 2019,

pour les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations n'utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. Je suis conscient qu'on ouvre là un champ compliqué à gérer. Je retirerai donc cet amendement après avoir entendu l'avis de la commission.

loi entre en vigueur le 1 septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l'entrée en vigueur du même titre II, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ces dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks. » Ce qui est proposé, c'est que ces produits puissent être vendus et distribués jusqu'au 1 septembre 2021 : il y a donc bien une date butoir pour la vente des produits sous ancien étiquetage.

pour un rappel au règlement. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement porte sur la gestion du temps réservé à chaque groupe.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis son essor il y a deux siècles, l'industrie a joué un rôle capital dans le développement et la puissance économique de l'Europe. Pourtant, les États membres de l'Union européenne n'ont jamais réussi à s'entendre pour mettre en place une politique industrielle active. Les conséquences de cette carence sont connues sans soutien stratégique pour affronter la libéralisation des échanges et l'ouverture des frontières, des secteurs industriels entiers ont été démantelés. Dans les territoires les plus durement touchés, les populations fragilisées expriment aujourd'hui leur ressentiment face à une Europe qui n'a pas tenu sa promesse de prospérité et n'a pas su, ou pas voulu, enrayer le cycle de la désindustrialisation. Dans notre pays, l'hémorragie se poursuit. On ne compte plus les dossiers stratégiques sur lesquels l'absence de politique industrielle européenne se conjugue à l'incapacité du Gouvernement à écouter les acteurs de notre industrie. Alcatel-Lucent, ou l'abandon du marché des télécoms : 400 emplois sacrifiés ; Ford, qui a vu son projet de reprise de l'usine de Blanquefort rejeté : 850 emplois ; Ascoval, ou l'abandon des matières premières : 300 emplois ; chez moi, en Seine-et-Marne, Arjowiggins, ou l'abandon de notre souveraineté pour les documents sécurisés : 240 emplois

Le Président de la République, qui n'hésite pas à brader les intérêts stratégiques de la France, ... Mais non ! ... notamment en matière agricole, a renoncé à toute ambition industrielle pour notre pays, mais s'est découvert une ambition pour l'industrie européenne. Espérons qu'elle ne connaisse pas le même sort que ses autres priorités européennes, lesquelles ont toutes, jusqu'à présent, été mises en échec : l'Union européenne ne peut pas se permettre de poursuivre sur la voie de l'indifférence industrielle. Face aux grandes mutations de l'économie mondiale, cette évolution ne peut mener qu'au déclassement industriel et, à terme, au déclin économique de la En effet, les pays émergents exercent une concurrence de plus en plus vive, y compris dans des secteurs où l'Europe pensait qu'elle aurait toujours une technologie d'avance. Par ailleurs, la révolution numérique et la marche vers la transition écologique se sont accélérées. Dans la course de vitesse qui s'est engagée pour dominer les nouvelles technologies et les nouveaux marchés qui en découlent, les entreprises américaines et chinoises ont clairement pris une, voire plusieurs longueurs d'avance. Enfin, l'ordre économique international est devenu dysfonctionnel. Les guerres commerciales amorcées par les États-Unis contribuent à le déstabiliser pis, les règles multilatérales sont de moins en moins respectées, à part peut-être par les Européens. La Commission et les États doivent prendre la mesure du bouleversement en cours et dépasser leurs réticences respectives pour élaborer enfin une stratégie industrielle européenne digne Les financements publics en faveur de la recherche devront non seulement être massifs, mais porter bien davantage sur les stades ultérieurs de l'innovation, jusqu'au déploiement industriel. Ils devront également s'accompagner d'une mobilisation plus importante qu'aujourd'hui des capitaux privés, notamment le capital-risque. Surtout, les actions de la Commission et des États devront être mieux coordonnées, soit par de grands programmes mobilisateurs favorisant les coopérations industrielles, soit par l'animation de pôles d'excellence technologique et industrielle. Une fois ce cadre établi, les autres politiques de l'Union européenne devront être mises en cohérence avec la priorité industrielle. l'a une nouvelle fois prouvé : le droit de la concurrence est concerné au premier chef, et il est indispensable de faire évoluer son application pour qu'elle soit plus en phase avec les réalités de l'économie contemporaine.

également comprendre que la consolidation et le rattrapage technologique des entreprises étrangères sont aujourd'hui beaucoup plus rapides qu'hier ; dès lors, elles peuvent conquérir des marchés sur lesquels les industries européennes détenaient peu de temps avant un avantage concurrentiel certain. La logique des régimes d'exemption par catégorie et des projets industriels d'intérêt européen commun pourrait également être élargie pour favoriser la formation d'une politique industrielle. Les secteurs définis comme stratégiques devraient ainsi bénéficier de règles dérogatoires assouplies, tant dans le domaine des aides d'État que dans celui des concentrations.

cette logique atteint aujourd'hui ses limites. Il faut désormais donner au projet européen une orientation plus offensive et plus protectrice, face à des concurrents qui ne jouent pas selon les mêmes règles.

Mais c'est également vrai de nos autres partenaires commerciaux, qui pour la plupart protègent leurs marchés et leurs entreprises tout en appliquant des normes bien moins strictes que les nôtres. L'Europe doit donc d'urgence imposer une plus grande réciprocité des échanges et renforcer ses outils de défense commerciale. D'ailleurs, elle a récemment amélioré ses instruments antidumping, et elle a élaboré de nouvelles règles pour le contrôle des investissements étrangers. C'est un pas dans la bonne direction, mais il faut aller plus loin. Ainsi, n'hésitons pas à mettre en place une taxation du carbone aux frontières de l'Europe ; renforçons massivement le contrôle des produits importés pour vérifier leur conformité aux règles d'accès au marché unique, qui est loin d'être toujours satisfaisante. L'adoption d'un instrument international sur les marchés publics doit également être une priorité. Un tel outil permettrait de restreindre l'accès des entreprises étrangères à nos marchés publics si leurs États usent, dans leurs propres marchés publics, de pratiques discriminatoires envers les entreprises européennes. Cette logique devrait même être amplifiée, s'étendre à tous les marchés, publics ou non, voire être complétée si nécessaire par un renouant avec le principe de préférence communautaire et réservant une part de la commande publique aux entreprises européennes, en particulier dans les activités dites « de souveraineté », comme la défense, l'aéronautique, l'énergie et les télécommunications. Il s'agirait d'un d'un pas décisif vers une véritable protection de nos technologies et de nos infrastructures critiques, qui sont par ailleurs de plus en plus liées aux infrastructures numériques et donc de plus en plus vulnérables face au pillage, à l'espionnage et au sabotage.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Cuypers, permettez-moi de vous dire avec quel plaisir je prends part à ce débat. S'il y a bien une conviction qui ne m'a jamais quittée, comme ancienne cadre exécutive d'entreprise industrielle et comme secrétaire d'État, c'est bien que le succès industriel français

une simple et bonne raison : face à la concurrence américaine ou chinoise, les bonnes réponses doivent être apportées au niveau continental. Cela n'aura échappé à personne : depuis quelques années, le paysage économique mondial a changé.

Face à ces menaces, l'Europe n'est pas restée les bras ballants. Nous avons su répondre de façon efficace, car unie, à la crise de l'acier, déclenchée par les importations massives d'acier en Europe. Nous avons modernisé nos instruments de défense commerciale pour mieux protéger nos entreprises face à une concurrence déloyale. Nous avons désormais un mécanisme européen de, ou de revue, pour contrôler les investissements étrangers en Europe dans les domaines stratégiques.

Les stratégies de ces pays sont assumées, globales, et bénéficient d'un soutien public ambitieux. À mon sens, l'Europe doit, elle aussi, être en mesure de proposer une stratégie ambitieuse, visible, centrée sur ses industries stratégiques.

le Conseil européen des 21 et 22 mars a appelé la future Commission européenne à mettre en place une stratégie industrielle dès la fin de l'année 2019. L'Allemagne et la France sont les moteurs de cette nouvelle politique. En Allemagne, Peter Altmaier a présenté une stratégie de politique industrielle qui marque une rupture forte par rapport à l'ordo-libéralisme traditionnel allemand. nos deux pays ont signé un manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXI siècle. Ce texte traduit une ambition commune pour faire de l'Europe un continent doté d'une industrie forte, à la pointe de l'innovation, capable de favoriser l'émergence d'acteurs d'envergure internationale. Avec les élections européennes et la constitution de la future Commission, Produire en Europe, avec de l'innovation européenne, des usines en Europe et des travailleurs européens, c'est possible ; c'est même encore plus possible avec la transformation technologique, qui nous permet de relocaliser de manière compétitive certaines productions en Europe. Mais, pour cela, il nous faut une impulsion politique nouvelle, autour de trois axes. Le premier axe consiste à armer nos entreprises face à la concurrence mondiale. Face à un protectionnisme américain assumé, face aux stratégies commerciales agressives de la Chine, l'Europe ne doit pas seulement être le bon élève du commerce international. Il nous faut renforcer drastiquement l'arsenal de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour le contrôle des subventions industrielles et le respect des règles de protection de la propriété intellectuelle.

d'ailleurs dit vous-même. Enfin, pour armer nos entreprises face à la concurrence mondiale, il est parfois nécessaire de constituer de grands groupes industriels. Pour que le refus de la fusion Alstom-Siemens ne se reproduise pas, les règles européennes de concurrence doivent évoluer. Sur certains marchés, peu nombreux et bien identifiés, il n'y a probablement pas de place pour plusieurs acteurs européens capables de concurrencer les acteurs américains, chinois ou indiens présents à l'échelle mondiale, qui sont souvent largement subventionnés ou qui bénéficient de marchés protégés. consiste à soutenir massivement l'innovation et son déploiement industriel sur le sol européen. Il faut tout d'abord coordonner nos efforts sur les chaînes de valeur stratégiques pour l'Union européenne- déterminées

Nous travaillons maintenant à un projet industriel avec l'Allemagne et d'autres partenaires pour produire en Europe des cellules de batteries électriques, composant indispensable à l'autonomie européenne sur les véhicules électriques.

Enfin, l'Union européenne doit davantage financer l'innovation de rupture, pour que l'Europe soit la première sur les sauts technologiques. Il est également primordial de créer une véritable union des marchés de capitaux, pour rattraper notre retard sur le capital-risque. enfin, s'attache à accélérer la transformation numérique et la transition écologique et énergétique de tous les secteurs industriels. Il n'y aura pas d'industrie forte en Europe sans une réponse complète et coordonnée à ces deux défis. Notre autonomie technologique et stratégique est en jeu. L'Union européenne doit garder la maîtrise de ces technologies clés en favorisant l'émergence d'acteurs de référence au niveau mondial en matière d'intelligence artificielle, de calcul quantique, d'internet des objets ou de. Nous n'avons pas à rougir des grands groupes européens en la matière, il nous faut combler notre retard technologique en soutenant le développement industriel de notre propre offre numérique souveraine. La lutte contre le changement climatique représente un coût pour nos sociétés et pour notre industrie, mais c'est aussi une chance, si on si on s'en donne les moyens, de positionner cette dernière à l'avant-garde mondiale et de gagner de nouveaux marchés. L'Europe doit focaliser ses financements sur le développement des technologies bas carbone et orienter les financements privés pour que l'industrie réalise les investissements nécessaires à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Il nous faut donc préserver la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale en adoptant des mesures de lutte contre les risques de fuite de carbone et en mettant en place un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Union pour des secteurs pilotes.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

je vous livre deux citations : « Nous voulons enfin prendre l'opportunité de développer la productivité, l'expansion de notre économie. » « Il faut une nouvelle approche de la politique industrielle en Europe.

que c'est enfin le moment de l'industrie en Europe, mais cela fait soixante ans que l'Union européenne suit une stratégie de mise en concurrence et de compétitivité des prix, une stratégie de refus de tout soutien public, d'affaiblissement des protections sociales, tournée vers la profitabilité des grands groupes au détriment du maillage territorial, une Les chiffres ne mentent pas : en plus de vingt ans, l'emploi industriel a reculé de près de 26 %, alors cessons les grandes déclarations Au-delà des chiffres, ce sont les emplois induits, les réseaux de PME, l'aménagement du territoire, les conditions de vie qui se dégradent. Ce sont des métiers, des fiertés ouvrières, qui disparaissent. Face aux défis de la révolution numérique, à la montée en puissance de la Chine, les propositions de la Commission et du Gouvernement ne remettent pas en cause une stratégie qui a pourtant échoué. Madame la secrétaire d'État, je ne suis pas garagiste, mais je sais que, lorsqu'un moteur est défectueux, refaire la carrosserie ne sert à rien ! Alors, faisons de véritables propositions, en rupture avec les précédentes. Dans cette perspective, mes questions seront les suivantes. Madame la secrétaire d'État, êtes-vous prête à soutenir l'idée d'un fonds d'investissement important à l'échelle européenne ? Êtes-vous prête à défendre nos marchés en imposant des visas écologiques et sociaux aux importations aux frontières de l'Union européenne ?

Madame la sénatrice Gréaume, vous indiquez que l'Europe avait pris en 1960 des positions très fortes sur l'industrie. Je crois me souvenir que, dans les années 1960 et 1970, elle avait effectivement une industrie particulièrement puissante au plan mondial. On ne peut donc pas dire que le marché européen a été un échec, bien au contraire. Nous, nous parlons des vingt dernières années. Je vous rejoins sur le diagnostic, il correspond d'ailleurs, au terme près, à celui que je viens de faire à la tribune. S'agissant des propositions que vous avancez,

la liste des entreprises qui licencient ou qui ferment ne cesse de s'allonger, certaines passent sous contrôle étranger, Saint-Gobain Pont-à-Mousson en est le dernier exemple. Face à la Chine et à l'Amérique, face à leur agressivité commerciale, il est urgent de refonder une politique industrielle européenne et de mettre en place une politique industrielle française, qui nous fait cruellement défaut. Il faut en finir avec la naïveté face aux grandes puissances, nous ne sommes pas seulement un continent de consommateurs, mais aussi un continent de producteurs. L'Europe ne doit être ni fermée ni offerte, les règles du jeu doivent être équitables, elles ne le sont pas : il n'y a pas réciprocité dans les échanges.

l'Europe sans industrie sera un continent faible, uniquement un marché. Refonder une politique européenne, c'est revoir les règles de la concurrence,

oeuvre une véritable politique commerciale et des investissements européens. Quelle est votre politique dans ce domaine et quelles sont vos orientations ? La parole est

Vous évoquez les problèmes de réciprocité, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour cela que nous avons réagi sur l'acier et que nous mettons en place des accords de libre-échange contenant les notions de réciprocité et d'ouverture sur les marchés publics. J'en veux pour preuve l'accord avec le Japon, qui vient d'entrer en vigueur. C'est pour cela, aussi, que nous entendons réviser les règles de la concurrence, vous connaissez notre point de vue sur le sujet. Il s'agit, d'abord, de définir le marché pertinent pertinent pour apprécier la concurrence qui s'exerce lors d'une consolidation : ce n'est plus le marché européen, mais le marché mondial ... Exactement ! C'est une réalité que nous vivons tous. Il faut également apprécier le marché avec une vision dynamique. Si l'on prend les parts de marché du passé, alors que les marchés peuvent se recomposer en cinq ans, et si l'on ne tient pas compte des appels d'offres à venir et de la réalité de la concurrence que ceux-ci suscitent, alors on est à côté de la plaque. C'est très exactement

Enfin, contrôler les investissements, cela correspond précisément aux décisions qui viennent d'être prises et que je mentionnais à la tribune, relatives au mécanisme de des investissements étrangers en Europe.

avait promis un plan industriel, il n'y en a toujours pas, mais il y a eu 110 licenciements ! Nous avons besoin d'un État stratège, qui nous fait cruellement défaut. Concernant Alstom, mettrez-vous en place une stratégie française à la suite de l'échec de l'absorption par Siemens ?

du Gouvernement. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez. Notre tissu industriel souffre, c'est un fait. Si je me félicite, en tant que parlementaire des Hauts-de-France, qu'une solution semble avoir été trouvée pour l'usine Ascoval, je ne peux que déplorer le sort réservé aux salariés d'Arjowiggins et je reste inquiet pour Arc International. Plus que jamais, nous devons soutenir nos entreprises en difficultés et, surtout, trouver de nouveaux axes de développement industriel. Les énergies nouvelles en font incontestablement partie. Pour résister à la mondialisation et à la concurrence des grandes puissantes émergentes, nous devons unir nos forces avec nos voisins européens, l'indique la récente déclaration commune de la France et de l'Allemagne publiée le 19 février 2019 et appelant à une véritable politique industrielle européenne. Nos deux pays ont d'ailleurs validé, à la fin de 2018, une feuille de route pour la création d'une filière européenne de la batterie de stockage d'énergie, ainsi que vous l'avez rappelé, madame Cette filière ambitionne d'accompagner la transformation de nos parcs automobiles avec un recours croissant aux véhicules électriques et hybrides. Ces batteries contribueront, par ailleurs, à l'alimentation en énergie de nos habitations. Pour y parvenir, il est vital que les constructeurs automobiles européens jouent le jeu et que l'Europe réponde présent en renforçant ses investissements dans le secteur privé, ce que rendra possible la reconnaissance de cette filière comme projet commun prioritaire d'investissements. Nos gouvernements espèrent obtenir ce label dès le premier semestre 2019, mais peut-être est-il déjà trop tard. Je fais référence à la construction en cours, en Allemagne, de la plus grande usine de batteries pour véhicules électriques. Un projet porté par la Chine Alors que l'Europe commence à réfléchir aux initiatives à reconnaître d'intérêt commun, la Chine monte les murs d'une unité de production de 55 hectares, investit 240 millions d'euros et crée 600 emplois avec l'objectif d'équiper 300 000 véhicules de marques allemandes et européennes. En résumé, nous sommes à nouveau très en retard, voire à la traîne. Alors que se profilent les élections européennes, n'est-il pas temps d'inventer une Europe réactive et efficace, capable de prendre des décisions aussi importantes que le soutien à une filière d'avenir ? Aujourd'hui, les processus décisionnels et l'absence d'harmonisation de nos cadres nationaux condamnent toute initiative de ce type et le résultat est devant nous : nos concurrents avancent bien plus vite et continuent de grignoter des parts de marchés là où nous devrions être en pointe. La parole

Par ailleurs, j'aimerais que l'on célèbre également les succès : Toyota investit 300 millions d'euros dans l'industrie automobile, AstraZeneca investit plus de 100 millions d'euros dans l'industrie pharmaceutique dans les Hauts-de-France, pour ne prendre que ces deux exemples.

d'améliorer la compétitivité de l'usine. Nous sommes donc plutôt confiants sur la situation de cette entreprise.

l'Europe se prive du bénéfice d'un marché plus large que ceux des États-Unis et de la Chine à cause de l'hétérogénéité de ses réglementations et de ses politiques, notamment en matière industrielle. Ainsi, dès avant le Brexit, et plus encore maintenant, le Royaume-Uni, traditionnellement peu interventionniste, affirmait néanmoins vouloir soutenir son industrie. L'Allemagne a été ébranlée par le rachat d'entreprises par de grands groupes chinois, sans que sa législation lui permette de s'y opposer. Une politique commune ou une convergence des règles est nécessaire, à l'instar de ce qui a été fait, avec succès, pour la plupart des réglementations sur les produits. Il est cependant un domaine dans lequel l'Europe a mis en place une politique commune : la concurrence. Je ne reviendrai pas sur la triste affaire Alstom-Siemens, déjà largement évoquée, mais, alors mais, alors que les consommateurs européens peuvent acheter des produits fabriqués dans le monde entier, cette politique empêche l'émergence d'acteurs européens puissants, sans grand bénéfice pour le consommateur et avec des dommages importants pour le tissu industriel du continent. votre prédécesseur l'avait justement dit ici même, nous ne pouvons pas faire reproche à Mme Vestager d'appliquer les textes, mais cela signifie donc que ce sont les textes eux-mêmes qu'il convient d'adapter. Madame la secrétaire d'État, que compte faire la France dans le cadre de la nouvelle Commission pour que les politiques industrielles des États membres soient mieux harmonisées entre elles et que l'on ne leur oppose plus

et ne bénéficie pas aussi facilement d'un tel avantage. Vous avez également mentionné les achats qui ont probablement fait bouger les positions allemandes sur l'ordo-libéralisme, notamment Kuka, une société de robotique extrêmement

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous débattons ce soir de la politique industrielle européenne. Je salue l'initiative du groupe Les Républicains qui a placé ce sujet essentiel au coeur de nos réflexions, quelques semaines avant les échéances que nous savons. Ce débat intervient aussi, et surtout, quelques semaines après un événement majeur pour l'industrie de notre continent : la Commission européenne a bloqué, début février, le projet de fusion entre Alstom et Siemens, tuant dans l'oeuf l'émergence d'un nouveau champion européen. Selon Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, cette décision se justifie, car « cette concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse. » Ces arguments ne sont pas à la hauteur des enjeux, ils révèlent l'absence criante, à Bruxelles, de vision politique claire en matière de stratégie industrielle. Il ne s'agit pas de remettre en question le principe de libre concurrence au sein du marché unique, mais simplement d'accepter la réalité d'un monde nouveau dans lequel les positions dominantes des entreprises européennes ne s'apprécient plus au niveau du marché unique, mais de la concurrence internationale. Pour que l'industrie continue d'exister sur notre continent, nous aurons besoin de champions européens qui puissent tenir tête à leurs concurrents américains et chinois. Dans quel périmètre le droit européen de la concurrence devra-t-il s'appliquer demain ? Quelles règles permettront de donner corps au principe de réciprocité ? Quelles actions le Gouvernement entend-il mener pour concilier, au niveau européen, respect de la concurrence et défense de nos intérêts continentaux ? La parole est

égal avec ses grands compétiteurs internationaux. Il nous aurait probablement permis, également, de concentrer l'innovation et de nourrir de nouvelles avancées technologiques susceptibles de donner ce quart d'heure d'avance stratégique qui fait la compétitivité d'une entreprise.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État. Il me semble que nous devrions nous en tenir à un principe clair de réciprocité avec nos partenaires commerciaux. Il y va de notre capacité à rester maîtres de notre destin industriel, en faisant le choix d'une économie qui reflète les valeurs fondatrices de l'Union européenne face aux géants étrangers d'aujourd'hui et de demain.

Son déploiement est un enjeu crucial pour nos opérateurs économiques comme pour nos concitoyens. Il ne s'agit pas, en effet, d'une simple amélioration technologique, mais d'une véritable révolution au coeur du monde ultra-connecté de demain.

le déploiement massif de flottes de voitures autonomes, ou encore le développement de « villes intelligentes » qui optimiseront leurs réseaux d'énergie ou de transport. On le voit, cette technologie est au coeur de l'industrie et de l'économie du XXI siècle. Le réseau 5G est déjà actif en Corée du Sud, il est en cours de déploiement aux États-Unis et devrait l'être en Europe en 2020. Pourtant, les Européens sont en train de prendre du retard en la matière, principalement en raison des enjeux de sécurité attachés à cette technologie, alors que deux de ses principaux acteurs sont chinois. En raison des transferts massifs de données inhérents à la 5G, la question de sa sécurité est en effet posée. Dans plusieurs pays européens, dont la France, des tests sont en cours. Cette question est cruciale, qu'il s'agisse de la sécurité des données à caractère personnel, de la protection des secrets de fabrication ou des secrets d'affaires, ou encore de la sécurité en matière de défense.

sont envisagées pour sécuriser le stockage des données ? Quant à la sécurité des données commerciales, industrielles ou miliaires, quelles sont les garanties exigées des fournisseurs d'infrastructures, du point de vue technique comme juridique ? Comment la France et, au-delà, l'Union européenne entendent-elles préparer cette étape aussi cruciale qu'urgente ? Pouvez-vous, enfin, nous confirmer qu'un déploiement en 2020 est toujours d'actualité ?

5G eux-mêmes, comme vous le savez, nous sommes en train d'en débattre en ce moment même à l'Assemblée nationale et vous aurez donc l'opportunité de discuter ce texte, qui vise à prévoir un dispositif permettant au Premier ministre d'autoriser spécifiquement

Dans ce manifeste, Paris et Berlin proposent que le Conseil européen bénéficie d'un droit de recours en vue de revenir sur les décisions de la Commission en matière de concurrence.

J'ai compris que Mme Vestager était plutôt ouverte sur le sujet. Je proposerai pour ma part que la Commission prenne en compte dans son appréciation l'ensemble du marché européen et réalise ses études et projections à moyen et long terme.

d'abord, l'évolution de l'économie mondiale et de ses zones de croissance nous force à constater que les bases de la politique de concurrence en Europe sont caduques aujourd'hui. Seront-elles revues avec le concours, le cas échéant, des règles et des sanctions extraterritoriales, qui me semblent être la seule solution

est à M. Jean-François Longeot. Madame la secrétaire d'État, parmi les trois dimensions de la politique industrielle européenne, le contrôle des concentrations, l'interdiction des aides publiques, et la répression des ententes et abus de domination, ce sont les deux premières qui recueillent sans aucun doute les critiques les plus virulentes. Si l'existence d'une politique européenne de concurrence a puissamment contribué à l'intégration économique européenne, celle-ci se voit désormais adresser bon nombre de reproches, qui devraient conduire l'Union européenne à s'interroger sur les évolutions à y apporter. Une fois de plus, l'histoire se répète avec Alstom. Après l'échec du rapprochement entre Aérospatiale, Alenia et De Havilland, le refus de l'accord entre Pechiney, Alcan et Algroup ou encore celui de la fusion Schneider-Legrand, sommes-nous condamnés à ne pas voir émerger de géants industriels européens dans les années à venir ?

-redoutent d'engager plusieurs mois de négociation avec la Commission européenne et, d'autre part, en raison de politiques industrielles nationales cloisonnées. Il est pourtant essentiel de défendre l'application du principe de réciprocité dans la compétition mondiale.

Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous présenter les mesures que vous comptez défendre dans ce domaine ? Après la politique agricole commune, comment mettre en place une politique industrielle européenne, que Nathalie Loiseau appelait d'ailleurs de ses voeux la semaine dernière ? La parole est à Mme la secrétaire

Concernant les règles de concurrence et notamment l'instance d'appel politique, l'une de nos propositions est de suggérer que le Conseil européen

ses marchés et ses entreprises. Si le débat sur les outils de défense commerciale reste animé, voire houleux, il n'est heureusement plus tabou. Il reste cependant un point sur lequel aucune riposte efficace n'a encore pu être élaborée, c'est l'extraterritorialité du droit américain, pratique qui s'apparente davantage à un racket organisé qu'a une simple distorsion de concurrence, puisqu'elle instrumentalise le droit pour déstabiliser, fragiliser ou placer sous surveillance les concurrents des entreprises américaines. Très juste ! En décembre dernier, on apprenait qu'Airbus risquait d'en être la prochaine victime. En plus d'une colossale amende, le groupe pourrait ainsi se voir couper l'accès aux marchés internationaux libellés en dollars. Il s'agirait d'une catastrophe qui laisserait le champ totalement libre à Boeing.

la plupart industrielles. Même si cela risque de changer avec Huawei, aucune entreprise chinoise n'a encore été visée, car l'administration américaine sait que Pékin n'hésitera pas à répliquer en s'en prenant aux sociétés américaines. Cette dissuasion, l'Europe n'est jamais parvenue à l'instaurer. L'activation du règlement dit « de blocage » de 1996 et le lancement du dispositif Instex- -en début d'année ont le mérite d'exister. ils restent largement inopérants, car ils ne sont pas sous-tendus par une volonté politique de ne rien céder face à la prédation américaine. Madame la secrétaire d'État, ma question est simple quelle stratégie crédible et efficace la France pourrait-elle proposer pour que l'Europe ne soit plus soumise aux injonctions américaines et qu'elle protège mieux son industrie des appétits de Washington ? La parole

1 avril. Ce mécanisme vise à surveiller l'impact des acquisitions d'entreprises ou de technologies stratégiques en Europe par des groupes étrangers. Il s'agit d'un premier pas en matière de défense commerciale de notre patrimoine industriel et technologique, bien nécessaire dans le nouveau contexte Un rapport récent de la Commission européenne sur les investissements directs étrangers montre que le poids prépondérant des investisseurs étrangers historiques en Europe, au premier rang desquels les États-Unis, tend à diminuer en faveur notamment de la Chine. Or la problématique essentielle pour les États-Unis était et reste celle des barrières douanières commerciales. En revanche, la Chine est bien plus intéressée par les technologies que nous développons en Europe, notamment en matière d'industrie aéronautique et de machines spécialisées, dernières années, l'Union européenne s'est certes dotée d'outils visant à améliorer sa capacité à résister aux offensives commerciales chinoises, mais l'action coordonnée des Européens doit être renforcée. Je pense en particulier au projet des nouvelles routes de la soie ou à la fragilité de certains États membres comme la Grèce, face aux investissements chinois, en raison de la perte de leur propre capacité industrielle. Aussi, le mécanisme de filtrage des investissements reste insuffisant face à ces enjeux. Il met en place un dispositif utile de coopération entre États, qui permettra un échange d'informations sur les filtrages en cours. En revanche, le texte adopté n'oblige pas les États à opérer ce filtrage et précise clairement que la décision d'approuver un investissement reste exclusivement du ressort national. La Commission européenne aura simplement la possibilité d'émettre une opinion. Il demeure donc indispensable de s'organiser, à la fois pour la protection des industries européennes et pour un meilleur encadrement des investissements étrangers dans les États membres tentés par des investissements chinois massifs.

je ne crois pas que les gouvernements européens versent dans la naïveté par rapport aux investisseurs étrangers. La situation a beaucoup évolué.

Segouin. Nous avons bâti l'Europe avec l'idée que l'union était indispensable pour faire face aux puissants que sont les États-Unis ou la Chine. C'était plutôt bien parti avec le marché commun et la monnaie unique, qui ont facilité la vie des entreprises. Mais, nous sommes loin d'en avoir fini. Chaque jour, en Chaque jour, en effet, nous constatons des différences réglementaires et politiques entre les États membres de l'Union européenne. Ces différences créent des concurrences toxiques et rendent difficile la production dans des domaines complexes et innovants. Nous sommes loin des produits. Je suis Je suis convaincu que nous pourrions conduire une politique commune avec, d'un côté, la convergence de certaines règles sur des chantiers majeurs et, de l'autre, des règles spécifiques pour que chaque État conserve ses caractéristiques. Il suffit de bien définir les sujets. Je pense par exemple à la lutte contre le réchauffement climatique. Imposer une taxe carbone sur les produits importés pour rendre compétitifs les produits fabriqués en Europe, c'est un chantier qui doit être suivi au sein de l'Europe et qui sera une juste réplique aux taxations appliquées par nos concurrents, comme la Chine ou les États-Unis.

France, l'imposition est trop forte, le coût du travail est trop cher et nos réglementations sont trop strictes. Bilan : les entreprises françaises n'ont plus assez de marges et deviennent vulnérables à chaque transmission. On a encore pu le constater le week-end dernier. Cette concurrence entre États bloque les rapprochements industriels et empêche l'émergence d'acteurs européens puissants, sans grand bénéfice pour les consommateurs. Posons-nous les bonnes questions : pourquoi ne fabriquons-nous pas de smartphone européen ? Pourquoi n'avons-nous pas de concurrent européen face à Amazon, Facebook ou Huawei,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la Cour des comptes a estimé récemment que la fusée Ariane 6 était trop conventionnelle pour faire de l'ombre à son grand rival américain SpaceX. Comme vous le savez, l'année 2019 est une année de transition entre Ariane 5 et le nouveau lanceur Ariane 6, dont le premier vol devrait intervenir dans le courant du second semestre de 2020. Il est donc impératif de poursuivre, voire d'amplifier les programmes de recherche, car Ariane 6 va arriver sur le marché mondial dans un environnement très concurrentiel. L'option de lanceurs récupérables doit faire l'objet d'études complémentaires en vue d'améliorer ses performances et de mesurer sa viabilité. Si on peut légitimement s'interroger sur les choix technologiques effectués par la filière européenne, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, qui nécessite une vision stratégique claire. nous a fait défaut ces dernières années, puisque Arianespace a perdu sa place de leader mondial de l'accès à l'espace commercial Dans ce contexte, j'aurais souhaité attirer votre attention sur l'absence d'une préférence européenne imposant aux États membres d'utiliser exclusivement le lanceur européen, contrairement à nos voisins américains, qui « lancent américain »,

gouvernementaux, militaires ou scientifiques -sera une réalité pour la fusée Ariane 6 ? La parole

on est tenté, soit de tout y mettre, soit de se concentrer sur un volet seulement, sur un concurrent en particulier ou sur un secteur. Ces différentes tentations illustrent le flou de ce qui constituerait une politique ou une stratégie industrielle, de surcroît européenne. Et derrière ce flou, se révèle un problème plus fondamental : nous ne serions pas capables, aujourd'hui, en 2019, en France et en Europe au moins, de déterminer la juste place et le rôle de la puissance publique, de l'État dans l'économie et dans la société. dans la société. Voilà quelques jours, à Hanovre, madame la secrétaire d'État, vous tweetiez qu'« une politique européenne, c'est mettre nos politiques de la concurrence, du commerce et de l'énergie au service de l'industrie Toutefois, vous ne précisez pas l'échelle la plus pertinente pour chaque volet et action de la politique industrielle. Vous évoquez, avec le ministre de l'économie et des finances, la constitution de « champions européens » ou de « géants européens capables de concurrencer les entreprises chinoises et américaines. Vous allez jusqu'à exprimer votre volonté de revoir les règles de la concurrence européenne, en particulier depuis le rejet, par la Commission, du projet de fusion

publié. Concrètement, comment concilier la constitution de géants avec la rigueur de notre administration européenne ? Dès lors, quelle place accordez-vous dans une politique industrielle européenne aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire ? La parole

ou, plus précisément, comme le montre le récent rapport sénatorial auquel j'ai pu participer, celui de la dépendance en principes actifs de l'Europe pour la fabrication des médicaments. découle une pénurie pour notre continent, qui se fait de plus en plus prégnante, représente un danger pour les malades et met en jeu notre sécurité sanitaire. Cette pénurie est en constante progression en France et en Europe depuis plusieurs années. sommes passés de 44 signalements de rupture de stock en 2008 à plus de 530 au 1 janvier 2019, pour une durée moyenne de quatorze semaines. Les chaînes de production pharmaceutique font face, de façon générale, à d'importantes problématiques, telles que les difficultés d'approvisionnement en matières premières par concentration des sites de production en principes actifs en Inde, Chine et Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les professionnels sont confrontés, en Europe, à une augmentation des coûts de production, parallèlement à des prix de vente de plus en plus contraints, les incitant à externaliser leurs outils de production européens vers des pays à main-d'oeuvre disponible, de bas coût et aux normes moindres. En 2018, l'Inde et la Chine concentraient 61 % des sites et 80 % des fabricants de substances actives des médicaments disponibles en Europe étaient situés en dehors de l'Union européenne, contre 20 % voilà trente ans. Il y a donc là une inquiétante perte d'indépendance sanitaire et l'urgence de mettre en place une véritable stratégie industrielle de relocalisation européenne de fabrication des principes actifs. L'Europe doit recréer les conditions d'une production de proximité et d'une filière « chimie » forte, afin de redémarrer la fabrication des médicaments d'intérêt vital actuellement importés et dont la livraison est irrégulière. C'est d'autant plus important que certains sites français, par exemple celui de Saint-Genis-Laval, dans le Rhône, sont menacés. Les sites de production chimique et pharmaceutique constituent un secteur particulier, auquel il est nécessaire d'appliquer des dérogations, en contrepartie, bien sûr, d'engagements.

Elle fournit un emploi à 35 millions de personnes et représente 20 % du PIB de notre continent. Depuis trente ans, son poids dans l'économie européenne n'a pourtant cessé de chuter. La concurrence des pays émergents, qui a fait tant de mal à nos industries traditionnelles, s'exerce maintenant de manière aussi pressante sur des secteurs à très haute valeur ajoutée, que l'on croyait pour longtemps à l'abri. Dans le même temps, des bouleversements technologiques majeurs rebattent avec une incroyable vitesse les cartes de la puissance industrielle, transformant des secteurs entiers aussi rapidement qu'ils créent de nouveaux marchés. L'organisation collective du commerce international est, quant à elle, en train de changer radicalement de nature. Ses règles multilatérales s'étiolent peu à peu dans la foulée du néoprotectionnisme américain et, surtout, de l'inexorable montée en puissance de la Chine, qui, rappelons-le, continue de profiter d'un traitement préférentiel lié à son statut d'économie en développement- ce qu'elle n'est plus -tout en réclamant les avantages liés au statut d'économie de marché- ce qu'elle n'est pas. La conquête du monde dans laquelle ce pays s'est lancé n'est donc pas alimentée uniquement par ses mérites propres, qui sont certes réels. Dans ce contexte, la nécessité de bâtir une politique industrielle à l'échelon européen apparaît, non plus comme une option, mais comme une obligation. La réalité économique ne laisse en effet plus guère le choix. Le premier axe est humain. L'industrie est et sera confrontée à un immense besoin de compétences, lié à l'évolution de ses métiers. Il est donc nécessaire que l'Union européenne soutienne les efforts d'investissements des États membres dans l'éducation, l'apprentissage et la formation professionnelle. Ensuite, un cadre stratégique de soutien au développement industriel doit être élaboré autour de l'identification des secteurs pouvant être qualifiés d'intérêt stratégique pour l'économie européenne. Dans ces domaines, la recherche et l'innovation devront être massivement soutenues, à la fois par des fonds publics en hausse et par une mobilisation accrue des financements privés, et les coopérations industrielles devront être facilitées et encouragées, notamment le lancement de grands projets structurants. Mais, pour que des leaders industriels européens, puis mondiaux, soient en capacité d'apparaître dans les secteurs prioritaires, la politique de concurrence devra opérer une importante évolution. Si l'on souhaite véritablement soutenir la réindustrialisation du continent, le droit de la concurrence devra également prendre en compte d'autres éléments que le seul intérêt du consommateur, notamment des impératifs tels que la préservation de l'indépendance technologique, de l'emploi ou des savoir-faire industriels. Enfin, si l'Europe s'est fondée sur les principes d'ouverture des marchés et de concurrence libre et non faussée, force est de constater que ces préceptes ne sont pas nécessairement ceux qui guident la politique économique du reste du monde. La définition d'une politique industrielle européenne n'ira donc pas sans une politique commerciale révisée sur le fondement d'une exigence de réciprocité des échanges. Instruments de défense antidumping et antisubventions, réciprocité des conditions d'accès aux marchés ou aux programmes de financements publics, contrôle renforcé des investissements étrangers dans les actifs stratégiques, meilleure vérification de la conformité des produits importés avec les règles européennes, tous ces thèmes sont aujourd'hui au coeur des discussions. Ils doivent trouver une concrétisation ambitieuse, et surtout efficace, pour que l'Europe s'affirme davantage dans la mondialisation. Sans stratégie volontariste, l'Europe industrielle risque de passer à côté des nombreux nouveaux marchés qui ne cessent d'éclore. Mais, ce faisant, elle risque surtout d'être balayée par des concurrents internationaux particulièrement déterminés et conquérants. Il est donc urgent de la réindustrialiser.

! Il ajoutait : « Elle y trouvera également le moyen de créer de véritables emplois, les emplois industriels étant un élément déterminant pour la création d'emplois de service nombreux. collègue, le contexte était alors favorable à ce que soit, enfin, forgée une politique industrielle et commerciale porteuse d'espoirs pour l'avenir. Nous étions en 1998 ! En ce domaine, on le voit, les rapports, communications, résolutions se sont succédé avec les mêmes constats, mais aucun n'a véritablement été suivi. Pourquoi en irait-il aujourd'hui différemment ? L'expression « politique industrielle » n'est plus un tabou. Une certaine prise de conscience semble enfin voir le jour, tant au niveau des institutions communautaires que des États membres, traditionnellement rétifs à une stratégie industrielle commune. Le manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXI siècle, publié le 19 février dernier, est un premier pas vers une vision stratégique de l'industrie européenne. C'est donc maintenant qu'il faut agir, pour permettre à l'industrie européenne de faire valoir pleinement ses nombreux atouts dans la compétition internationale. Nous en